période à Personne, sur nos travées, ne peut se satisfaire d'une situation dans laquelle la protection sociale des Français de l'étranger n'est acquise qu'après un délai de carence qui n'est imposé à aucun Français sur le territoire national.